Si le sujet est juridiquement complexe, pour parvenir à la fin de l'exonération de taxes énergétiques, d'autres voies existent, plus en phase avec une vision positive de l'écologie. Certaines compagnies les ont mises en oeuvre. J'en citerai quelques-unes : le système de, qui consiste à laver les fumées émises par les bateaux ; le passage du fioul lourd au gaz naturel liquéfié (GNL),

20 % ; l'utilisation d'une pile à combustible fonctionnant au GNL, qui permettrait de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux moteurs classiques.

Pour avoir, avec d'autres collègues, rencontré certains acteurs de la filière, je dois cependant signaler à notre assemblée certains retards d'infrastructures dans nos ports, encore trop faiblement équipés de dispositifs de fourniture électrique pour les navires.

Il est proposé que le bénéfice du taux réduit s'applique à l'ensemble de l'électricité utilisée pour le fonctionnement du site, au sens de l'arrêté préfectoral d'autorisation dudit site. Cette taxation réduite est justifiée par l'activité de ces installations dites « vertueuses qui s'inscrit pleinement dans la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement, et qui participe également au développement de l'économie circulaire et solidaire des territoires. Ces énergies vertes sont généralement consommées localement dans le cadre de projets globaux, en partenariat avec des collectivités territoriales ou des entreprises. Les gains dégagés par la réduction de TICFE permettraient de limiter les dépenses des collectivités locales pour la valorisation énergétique des déchets résiduels et soutiendraient les effets nécessaires à la mise en place du document européen de référence

moins 50 % lorsque le rendement énergétique est au moins égal à 65 % et moins 75 % lorsque le rendement énergétique est au moins égal à 70 % et que les déchets sont issus d'opérations de tri performantes.

ainsi libellé : La parole est à M. Jean Bizet. Conformément à l'article 256 A du code général des impôts, une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d'électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En pratique, la jurisprudence administrative présume qu'il n'y a pas de livraison, donc pas d'assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n'excède pas 3 quelle que soit la nature du contrat d'achat. Cette limite de puissance est exclusivement d'usage et n'apparaît nulle part dans le code des impôts, pas plus que dans le code de l'énergie. Par extension, la jurisprudence administrative a considéré que ce seuil de 3 kilowatts crête s'appliquait également à la TVA à percevoir dans le cadre de la pose et de la fourniture des équipements de production des installations de moins de 3 kilowatts crête, au sens de son application de l'article 279-0 du même code. Par extension, cette même jurisprudence considère que, pour les installations collectives, ce seuil est entendu par logement. L'objet du présent amendement est donc de mettre la législation fiscale en cohérence avec la réalité de la demande des citoyens et la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique, en proposant d'élever le seuil d'application du taux de 10 % de TVA de 3 à 9 kilowatts crête, et donc d'assujettir seulement

Notre collègue Jean Bizet nous dit que le seuil du non-assujettissement à la TVA pour les petites installations ne correspond plus à la réalité du marché. Il nous dit, sans doute à juste titre,

que le particulier consomme toute sa production sans la soumettre à la taxe. Il nous paraît difficile d'aller au-delà. En tout état de cause, je rappelle que le bénéfice de la franchise de TVA est acquis jusqu'à 82 800 euros

le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité́ permet aux États membres de prévoir des exonérations partielles ou totales des taxes sur l'électricité d'origine renouvelable. Il est proposé, au travers de cet amendement, de favoriser le développement de l'électricité renouvelable en exonérant de TICFE les opérations d'autoconsommation collective régies par l'article L. 315-2 du code de l'énergie. Quel est l'avis de la commission ?

messieurs les sénateurs, je voulais vous signaler que le Gouvernement n'est pas opposé par principe à un traitement fiscal spécifique de l'autoconsommation collective et que des discussions ont été engagées sur ce point avec les professionnels pour trouver le juste dispositif. Elles ne sont pas achevées à l'heure où je vous parle.

L'amendement tend également à supprimer la réduction forfaitaire de 1 centime d'euro par mégawattheure, qui ne serait plus justifiée, dans le cadre d'une exonération de TICGN pour le biogaz injecté dans le réseau. Dans un premier temps l'exonération devrait donc être neutre pour les recettes de l'État.

de TICGN le biogaz seulement s'il n'est pas mélangé avec du gaz naturel d'origine non renouvelable et à appliquer une réduction forfaitaire de 1 centime d'euro par mégawattheure sur le gaz mélangé à du biogaz, ce qui revient à taxer de façon identique le gaz fossile et le biogaz, dès lors qu'ils sont injectés dans le réseau. Ce faisant, il supprime l'incitation fiscale à développer l'usage du biogaz, puisque l'ensemble des consommateurs de gaz naturel bénéficient de cette réduction forfaitaire due à la présence de biogaz injecté dans le réseau, dès lors dénuée de sens. Le présent amendement vise à rétablir l'exonération de TICGN pour le biogaz injecté dans le réseau.

C'est pourquoi il est indispensable de rétablir l'exonération de TICGN, de façon à permettre la transition du gaz vers les énergies renouvelables. C'est une disposition indispensable pour contribuer à progresser vers une économie neutre en carbone. Le gaz renouvelable peut contribuer à réduire de 1,4 à 1,9 million de tonnes les émissions de CO2 à l'horizon 2023. La méthanisation est un modèle économique durable, qui, à travers les cultures dédiées, offre des débouchés économiques importants, notamment pour notre agriculture. De nombreuses collectivités se sont déjà lancées dans des projets en partenariat de transformation en biogaz.

Cette conversion réalisée par les services du ministère de la transition écologique et solidaire a été faite de manière à tenir compte de l'ensemble des spécificités du réseau d'approvisionnement en gaz naturel. En particulier, a bien été pris en compte l'approvisionnement en gaz B des stations, gaz naturel pour véhicules situés en région Hauts-de-France or le taux de conversion B diffère de celui du gaz H- je rentre dans les détails -, qui approvisionne l'ensemble des autres stations. Cette particularité explique les résultats différents qu'ont pu mettre en avant certains opérateurs.

de l'article 265 du code des douanes. Cette clarification a encore été réaffirmée par la loi relative à l'énergie et au climat, dans son article 50. La rédaction actuelle de l'article 17 remet en cause cette exonération totale en n'exonérant plus que la part de consommation de biogaz se rapportant à la production d'électricité, soit environ 50 %. Or la chaleur générée lors de la production d'électricité n'est pas systématiquement récupérée ou valorisée, dans la mesure où la production de chaleur fatale est inhérente à la production de biogaz, donc d'électricité. Lorsque la chaleur n'est pas récupérée, elle ne peut pas être assujettie à une taxe intérieure de consommation, car cela reviendrait à taxer les produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité,

exonéré dans les installations de cogénération, qu'il soit utilisé comme combustible- cogénération chaudière -ou comme carburant- cogénération moteur. Ces amendements identiques sont donc déjà satisfaits. Par ailleurs, avec la rédaction

ou dans les travaux ayant permis d'aboutir aux mécanismes de soutien à la production d'électricité renouvelable à partir de biogaz et que ce soit par les acteurs économiques ou par les autorités publiques, y compris la Commission de régulation de l'énergie (CRE). (CRE). Cette disposition est donc inapplicable aux installations de cogénération bénéficiant d'un tarif d'achat ou d'un complément de rémunération de l'électricité produite à partir de biogaz.

prioritairement au chauffage des serres maraîchères : il s'agirait d'aider financièrement la production sous serre de légumes de contre-saison, en particulier des tomates, à l'aide de chauffage au gaz naturel. Pour un hectare de serre chauffée, le remboursement annuel passerait de 6 666 euros à

plutôt que de soutenir des productions de contre-saison, il conviendrait d'accompagner le changement vers des modes de production vertueux sur le plan environnemental et de limiter la concurrence déloyale-

d'année en année. En outre, il convient de travailler à une véritable reterritorialisation de l'alimentation, notamment la restauration collective ou les projets alimentaires territoriaux. Ce faisant, on diminuera efficacement le recours aux importations et on garantira

qui broie nos agriculteurs. C'est important de le dire ! On parle beaucoup d'agri-bashing : l'agri-bashing, ce n'est pas ce que l'on veut faire croire. Qui défend les agriculteurs ? Qui défend l'agriculture ? Qui défend la ruralité ? Sont-ce ceux qui soutiennent la concentration et l'industrialisation agricoles ? Ma réponse est

dernière, le Sénat a déjà proposé de revoir les critères du malus, compte tenu notamment du caractère dynamique de ses recettes, signe, selon nous, que le calibrage n'était pas parfaitement adapté.

du mieux-disant environnemental ! Au lieu de cela, vous gardez les vieilles méthodes de l'écologie de rendement en drapant la hausse du malus d'un vert bien pâle et en le recouvrant d'un vernis bien fade.

contrevient à toutes les règles d'une bonne fiscalité écologique

si la logique environnementale est compréhensible, le palier défini est extrêmement haut, notamment pour les plus modestes.

Plus de sévérité pour les véhicules polluants : ainsi peut se résumer le nouveau malus automobile. L'adoption d'un nouveau protocole d'homologation a été l'occasion de réviser les barèmes et de pénaliser plus lourdement les acheteurs de voitures émettant beaucoup de CO2. Si cette logique environnementale et désincitative est compréhensible, le palier à franchir est extrêmement élevé, notamment pour les classes les moins aisées. Nous déplorons la tournure prend la prime à la conversion, révisée cet été, en parallèle du système de bonus-malus automobile. Ce dispositif a été réduit et la prime à la conversion, désormais restreinte à l'achat

Depuis 2017, des plafonds d'amortissement non déductibles sont appliqués en fonction des émissions de dioxyde de carbone des véhicules. Pour les véhicules à très faibles émissions, ce plafond de déduction fiscale est établi à 30 000 euros, contre 18 300 euros pour un véhicule thermique. Cependant, ce plafond n'est plus en adéquation avec le marché actuel des véhicules électriques. La diversification des modèles et les montées en gamme permettent maintenant aux entreprises de s'équiper de véhicules adaptés à leurs besoins. Cependant, les véhicules électriques présentent toujours un surcoût important et un coût total de possession défavorable par rapport à leurs équivalents thermiques. Cet amendement tend donc à relever le plafond applicable aux véhicules émettant moins de vingt grammes de dioxyde de carbone par kilomètre à 45 000 euros.

diminuer de 6 000 à 3 000 euros. Il s'agirait d'un signal très négatif qui aurait des répercussions importantes sur les ventes des véhicules. Dans ce cadre, il semble utile de faire évoluer le barème d'amortissement des véhicules électriques à batterie et à pile à combustible pour inciter à leur acquisition. À ce jour, le calcul de l'impôt sur ces véhicules ne prend pas en compte la fraction de leur prix d'acquisition, qui dépasse 30 000 euros. Cet amendement vise à porter ce plafond à 45 000 euros, afin d'augmenter les sommes pouvant être déduites des bénéfices industriels et commerciaux.

en portant le plafond du prix d'acquisition à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l'établissement de l'impôt de 30 000 à 33 000 euros pour les véhicules à très faibles émissions et de 20 300 à 24 300 euros pour les véhicules à faibles émissions. Il s'agit d'inciter fiscalement les entreprises à acquérir des véhicules électriques et hybrides afin d'accélérer le verdissement du parc automobile français et d'atteindre les objectifs de réduction

sur le principe des aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules d'origine fonctionnant au superéthanol E85. Le décret du 16 juillet 2019 établit pour les particuliers la prise en compte d'un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au superéthanol E85 afin de tenir compte des importantes réductions d'émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l'ensemble de son cycle de vie. Il s'agit donc d'un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d'égalité devant l'impôt, puisqu'il tend à harmoniser la règle appliquée, d'une part, aux citoyens, d'autre part,

de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) réduite, la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburant, l'exonération de la taxe sur les certificats d'immatriculation au profit des régions, la minoration du malus écologique et la prime à la conversion,

Par ailleurs, les véhicules fonctionnant au superéthanol bénéficient déjà d'un barème favorable au titre de la deuxième composante du tarif de la TVS, assise sur les émissions de polluants. De surcroît, les plafonds retenus dans les différents amendements pour exonérer les véhicules avant abattement de 40

Cet amendement vise à introduire un critère de poids dans le calcul du bonus-malus des véhicules automobiles. Le dispositif de malus existant n'est plus efficace, puisque, au cours des trois dernières années, les émissions de CO2 des véhicules neufs sont reparties à la hausse et que 90 % des véhicules vendus actuellement ne sont soumis à aucun malus ou sont soumis à un malus inférieur à 500 euros. Le projet de loi de finances ne prévoit qu'une évolution très limitée la hausse du barème pour calculer les émissions de CO2 des véhicules ne changera donc la donne qu'à la marge. La question du poids des véhicules ne peut plus être ignorée. Un récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie indique que les SUV aujourd'hui responsables de la deuxième plus forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, derrière le secteur de l'énergie. Introduire ce critère permettrait de mieux prendre en compte les externalités, notamment celles qui tiennent au cycle de vie du véhicule. Les ventes de SUV, ces véhicules 4x4 de ville, très dopées par la publicité, sont en train d'exploser et représentent aujourd'hui pratiquement 40 % du marché de l'automobile en France. Il s'agit de véhicules lourds, si bien que, en France comme dans le reste du monde, ils sont devenus l'un des

De plus, prendre pour critère le poids des véhicules permet de limiter les risques de fraude, car c'est un indicateur plus fiable que la mesure d'émission de CO2, qu'il complète. Nous proposons

Les émissions de CO2 sont calculées à l'échappement et non sur l'ensemble du cycle de vie. Or, plus un véhicule est lourd, plus il a un impact environnemental important à la fabrication. Si l'on veut réduire fortement les émissions de CO2 des voitures particulières, il est donc essentiel de réorienter le marché vers des voitures plus légères et moins émettrices.

d'une issue différente. Il s'agit d'enrichir le bonus-malus par un indicateur basé sur le poids du véhicule. Le malus comprendrait alors deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et la masse du véhicule. en compte du poids est essentielle pour lutter contre le développement des grosses voitures, qui ne répondent pas aux enjeux de transition écologique. En effet, et comme le souligne le très récent rapport de France Stratégie, les émissions de CO2 des voitures neuves dans les conditions de conduite réelles n'ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan est principalement la conséquence d'une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Pourtant, l'augmentation du poids des véhicules pose de sérieux problèmes, y compris pour les véhicules dits propres. En effet, elle entraîne, de fait, une augmentation de la consommation d'énergie. Par ailleurs, la production de ces grands véhicules est particulièrement consommatrice en ressources naturelles et en énergie, notamment lorsque d'imposantes batteries électriques sont nécessaires. Selon France Stratégie, un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu'une petite voiture essence.

WLTP. Initialement envisagé au 1 janvier 2020, le passage à la norme WLTP doit finalement être repoussé, le temps de mettre en place un nouveau certificat de conformité électronique. L'article 18 prévoit ainsi une entrée en vigueur à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1 juillet 2020. Par conséquent, le barème du malus applicable au 1 janvier 2020, qui est durci par rapport à celui de cette année, sera remplacé au cours du premier semestre 2020 par un nouveau barème. Or, bien qu'il s'applique à partir d'un niveau d'émissions plus élevé, ce nouveau barème ne permettra pas d'assurer la neutralité fiscale du changement de norme pour l'ensemble des véhicules. En effet, alors que, dans l'ancien système, la valeur des émissions était mesurée par familles de véhicules sur la base des émissions du véhicule représentatif de chaque famille le plus favorable, la norme WLTP conduit à attribuer un niveau d'émissions à chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques. Le passage en cours d'année au système WLTP conduira donc à une augmentation du montant du malus sur certains véhicules, ce qui sera source de complexité pour les professionnels comme pour les consommateurs, qui auront beaucoup de mal à s'y retrouver au moment d'acheter leurs véhicules.

particulier, il fusionne les deux taxes fixes à l'immatriculation. La délivrance du certificat d'immatriculation, communément appelé carte grise, est soumise au paiement d'une taxe dite régionale, à laquelle correspondent plusieurs cas d'exonération, selon le type de véhicule-

L'article 18 a notamment trait aux émissions de dioxyde de carbone, à la puissance fiscale pour charges de famille et à l'exonération de malus en raison d'invalidité. Ces dispositions s'appliquent en cas d'achat, de crédit-bail ou de location avec option d'achat, mais il semble que la location de longue durée n'ait pas été prise en compte, ce qui crée une distorsion entre les différents usages de la voiture.

À défaut de prise en compte d'une période minimale entre la première immatriculation du véhicule en France et la nouvelle immatriculation consécutive à sa transformation de véhicule professionnel en véhicule de tourisme, la mesure aurait un effet négatif

pour atteindre l'objectif fixé par l'Union européenne à l'horizon de 2020 et réaffirmé par le Gouvernement dans le plan Climat : un taux moyen d'émissions de CO2 de 95 grammes par kilomètre pour les voitures neuves vendues. est par ailleurs imposé aux constructeurs de voitures particulières neuves par le règlement européen. À l'heure où l'on constate que le transport est le seul secteur de l'Union européenne n'ayant pas enregistré de baisse notable des émissions de CO2 depuis 1990 et que la France, je le répète, est condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour son inaction en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, l'État se doit de maintenir la trajectoire pour atteindre l'objectif de 95 grammes de CO2 par kilomètre en 2020.

comme le ministre Bruno Le Maire l'a récemment envisagé dans la presse. Nous proposons ainsi que le tarif augmente de 500 euros par gramme de CO2 supplémentaire émis. L'amendement

Il est impératif de maintenir cet objectif pour le secteur automobile. En outre, l'amendement vise à déplafonner le malus à partir de 173 grammes de CO2 par kilomètre et à majorer le tarif applicable de 500 euros par gramme supplémentaire de CO2 émis. Le ministre de l'économie s'est montré favorable à une telle mesure,

Cet amendement vise à modifier une référence de date dans l'article 18. En effet, il est prévu que plusieurs dispositions du code général des impôts s'appliquent pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisés en vue de liquider

n° I-117 rectifié . Cet amendement vise à exonérer les véhicules privés professionnels de transport des personnes à mobilité réduite de la taxe sur les véhicules polluants. En effet, de nombreux établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif se sont dotés de véhicules adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite, mais ne peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur les véhicules polluants, qui ne concerne que les particuliers. L'extension de ce dispositif à une plus grande partie des véhicules carrosserie « handicap » permettrait aux établissements de réaliser des économies et de renouveler plus régulièrement leur parc automobile spécialisé.

que nous aurons à l'article 19 -de prolonger l'exonération, en vigueur depuis 2005, de taxe à l'essieu pour les véhicules utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre des travaux publics. Sont visées les grues installées sur un châssis routier ou encore les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier. Ces véhicules sont exonérés depuis 2005, mais cette exonération doit faire l'objet d'une décision de la Commission

: ... Ah ? ... augmenter la fiscalité écologique tout en diminuant les impôts qui pèsent sur la compétitivité des entreprises pour les inciter à relever les enjeux

alors que le trafic routier de marchandises en France est assuré par des poids lourds sous pavillon étranger à hauteur de 40 %. Le régime de la TSVR dégrade la compétitivité des entreprises françaises de transport de marchandises par rapport à leurs concurrents étrangers, dispensés de contribuer aux coûts d'entretien des infrastructures routières. Son coût de recouvrement est par ailleurs élevé.

de reprendre un dispositif existant. Depuis le Grenelle de l'environnement, les transporteurs sont contraints d'informer les chargeurs ou les donneurs d'ordre du coût carbone de leur transport.

les l'ouverture des Assises nationales de la mobilité, voilà plus de deux ans, une question fait débat : comment faire contribuer les poids lourds étrangers qui transitent par la France à l'entretien des infrastructures de transport ? L'une des pistes régulièrement évoquée par le Gouvernement aucours des derniers mois est la mise en place d'une vignette obligatoire pour les poids lourds. Or la solution finalement retenue à l'article 19, qui consiste à augmenter la taxe sur les carburants due par le transporteur routier de marchandises reposera

France. Par conséquent, ils continueront à utiliser et à dégrader les infrastructures sans contribuer à leur entretien. Il y a donc tromperie sur la marchandise. On peut également regretter que cette hausse de la fiscalité soit uniquement conçue dans une logique de rendement budgétaire à pallier le manque de moyens de l'État pour financer les infrastructures de transport et qu'elle ne s'inscrive pas dans une réflexion de plus long terme sur la transformation de ces secteurs pour les accompagner à réaliser leur transition énergétique en s'orientant vers des alternatives moins émettrices de gaz à effet de serre. C'est pourtant ce que demandent les transporteurs :avoir de la visibilité sur l'évolution du cadre fiscal et réglementaire, et bénéficier d'un accompagnement pour réduire leurs émissions de CO2 à travers un véritable contrat de filière. Le secteur a par ailleurs fait une proposition alternative intéressante, qui consiste à taxer les chargeurs qui recourent à une prestation de transport plutôt que les entreprises

en mettant en place une éco-contribution. Monsieur le secrétaire d'État, je vous poserai donc trois questions très simples. Pourquoi avoir renoncé à l'ambition de faire contribuer les poids lourds étrangers à l'entretien de nos infrastructures de transport ? Que répondez-vous aux transporteurs qui demandent de la visibilité et un accompagnement pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ? Pourquoi avoir refusé de reprendre leurs propositions alternatives visant àtaxer les chargeurs plutôt que les transporteurs ? La parole est à M. Olivier Jacquin,

pour tenter d'inscrire le secteur des transports dans la transition énergétique et dans le principe du pollueur-payeur. Le rapporteur Didier Mandelli, qui avait accompli par ailleurs un excellent travail,

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est presque minuit. Comme convenu avant la suspension, je propose de prolonger la séance afin d'achever l'examen des dispositions relatives à la fiscalité écologique, c'est-à-dire jusqu'à l'article 33 inclus.

que je gagnais suffisamment pour ne pas avoir grand-chose à faire d'une taxe complémentaire sur le diesel ou sur l'essence, puisque je prenais l'avion et que le kérosène n'était pas taxé.

l'équivalent de près de 50 % du prix d'un billet. Il pèse sur la compétitivité de nos compagnies aériennes et de nos hubs. [ ...] La [ ...] conviction que je voudrais partager, c'est que nous pouvons collectivement faire mieux pour la compétitivité économique de notre pavillon.

la transition écologique et le défi qui s'impose au secteur de l'aérien, vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur général, le renouvellement des flottes compte souvent pour beaucoup. Ainsi, Air France renouvellera 50 % de sa flotte d'ici à 2026.

Nous proposons en effet que cette taxe soit progressive selon le type de billet et frappe plus lourdement les billets de première classe ou de « », pour conjuguer l'exigence environnementale avec la justice sociale.

d'aménagement du territoire. En effet, les liaisons qui ne seront pas considérées par la Commission européenne comme soumises à une obligation de service public risquent de se voir appliquer la réglementation européenne relative aux aides d'État et, par conséquent, la présente hausse de taxe sur les billets d'avion. Afin d'éviter de faire courir un risque juridique à des liaisons qui jouent un rôle essentiel dans le désenclavement de certains territoires, les conditions d'entrée en vigueur de la hausse de taxe seront les mêmes pour tous les types de liaisons aériennes,

de la Commission européenne, mais c'est inutile : il n'y a pas de difficulté liée au régime des aides d'État, en vertu de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cet amendement tend à organiser la suppression de l'éco-contribution sur les billets d'avion une fois que l'Union européenne adoptera une taxe de même nature. Il est clair qu'il faut mettre en oeuvre une solution européenne coordonnée pour réduire les émissions de carbone

Si ce soutien à l'innovation technologique dans le domaine environnemental doit être soutenu, il faut aussi noter les limites de ce marché carbone. En effet, la volatilité des prix des ressources, d'une part, et l'interaction avec les autres politiques de l'énergie et du climat, d'autre part, rendent difficiles les projections sur ce fonds. Elles n'encouragent pas vraiment les États à mener une politique ambitieuse en matière de réduction de gaz à effet de serre. Néanmoins, dès lors que les produits des enchères sont affectés à cette politique publique, les membres du groupe socialiste et républicain soutiendront une telle mesure, tout en regrettant son manque d'ampleur.

! L'article 32 prévoit également que le montant de la taxe d'aménagement acquittée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes reversé au CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

relatives au bonus automobile et à la prime à la conversion au sein du budget général de l'État. Elle rendrait par conséquent beaucoup moins lisible la politique de soutien au renouvellement du parc automobile, en mettant fin à l'affectation directe de la recette du malus au soutien à l'acquisition de véhicules propres. Or le dispositif du bonus-malus ne fait sens que parce que les recettes du malus perçues pour les véhicules polluants sont directement affectées à l'achat de véhicules peu polluants. Je vous invite donc, mes chers collègues, à maintenir ce compte d'affectation spéciale,